Le dispositif proposé tend à instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement, pour des biens acquis entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

le respect des plafonds de loyer et de ressources en cas de mise en location. L’exonération est plafonnée à 150 000 euros par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.

de prélever certains biens déterminés composant la communauté tels qu’ils ont été énumérés dans le contrat de mariage ou dans le changement de régime matrimonial. Cette disposition est éminemment protectrice pour le conjoint survivant : premièrement, sa faculté de choix ne s’ouvre qu’au jour du décès, ce qui lui permet d’adapter sa décision en fonction des circonstances le jour dit ; deuxièmement, uniquement en présence d’enfants communs et comme tout avantage matrimonial, il n’est pas limité par la réserve des descendants. En outre, compte tenu de la facilité, désormais plus grande, très récemment donnée par la loi civile pour modifier le régime matrimonial, cette faculté est appelée à connaître un développement significatif. Depuis quelque temps, l’administration fiscale entend soumettre l’exercice de cette faculté par le survivant au droit de partage. Or, selon les termes mêmes du code civil, il s’agit d’un prélèvement « avant tout partage qui permet précisément à l’époux survivant d’éviter toute indivision avec ses cohéritiers. En l’absence d’indivision, il ne peut y avoir de partage et, en l’absence de partage, aucun droit proportionnel ne peut donc être perçu lors de l’exercice d’un préciput. Quel est l’avis de la commission ?

auteurs du présent amendement demandent une prorogation de l’exonération du droit de partage de biens héréditaires en vigueur jusqu’en 2027. Compte tenu des tensions qui existent sur le marché immobilier de l’île, il est indispensable de proroger ce dispositif qui va dans le sens du maintien du patrimoine par transmission au sein des familles.

n’entraîne une hausse des tarifs pratiqués par les entreprises du secteur concerné.

le bien transmis, serait accordée sous certaines conditions précisées dans le texte de cet amendement. En outre, pour être complet, ce dispositif doit être élargi à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.

avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement et signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires. De plus, une attestation de bonne exécution des obligations du contrat devra être fournie. Parmi nos

signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques. Je précise à mon tour qu’une attestation de bonne exécution des obligations du contrat devra être fournie.

d’instaurer une taxe de 1 % sur toutes les successions pour financer le déficit de plus en plus lourd de la branche autonomie, qui va passer de 6 milliards

de la fraction des parts ou des actions imposables comme pour celle des biens et droits immobiliers imposables, que les dettes contractées par le redevable et afférentes à des actifs imposables le soient directement ou par l’intermédiaire d’une société détenue par le redevable. Il prévoit à cette fin que, pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne soient pas prises en compte. Pour que l’imposition en résultant n’affecte pas la capacité contributive du redevable, il prévoit également que cette nouvelle règle ne doit pas avoir pour effet de porter la valeur des parts ou actions imposable à l’IFI, déterminée conformément au 2° de l’article 965 du code général des dans les conditions de droit commun. Afin de renforcer cet objectif d’égalité de traitement, le présent amendement tend à prévoir que la valeur imposable à l’IFI des droits sociaux résultant de l’exclusion des passifs

Le recul de la méthode scientifique implique de se fonder sur les 41 milliards d’euros de dividendes versés par les sociétés financières, nets de ceux qu’elles ont reçus.

Selon France Stratégie, « l’instauration du prélèvement forfaitaire unique n’a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l’investissement significativement différente de celle des autres ». a non pas davantage d’investissements économiques, mais davantage de dividendes distribués, ce qui engendre une inégalité entre fiscalité du travail et du capital, une inégalité en faveur

« Si vous avez des revenus élevés et que vous cherchez à réduire votre charge fiscale, la peut être une option attrayante. Cependant, si vous cherchez à soutenir un système plus équitable et à financer des programmes sociaux, préférez le barème progressif. Voilà ce que conseille leblogdudirigeant.com, que je remercie pour son pragmatisme sans appel ! Il y a donc deux mondes qui s’affrontent. Pour notre part, nous sommes de ceux qui souhaitent soutenir un monde équitable. C’est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, de mettre un terme au mécanisme de prélèvement forfaitaire unique.

Une étude réalisée par l’Institut des politiques publiques en 2023 montre que les soixante quinze foyers les plus riches du pays sont proportionnellement moins imposés que les autres contribuables. L’instauration de la et la suppression de l’ISF ont accentué cette tendance en diminuant la participation des plus riches à notre système de redistribution. La a été conçue de nos concitoyens qui ont les moyens financiers d’accéder à l’information nécessaire pour comprendre les règles fiscales. La combinaison du PFU et la réorganisation de l’impôt de solidarité sur la fortune ont des effets préjudiciables à moyen et à long terme sur nos finances publiques et sur les politiques qu’elles soutiennent.

C’est d’ailleurs l’une des recommandations du rapport des deux députés, Jean Paul Mattei – membre de la majorité présidentielle – et Nicolas Sansu. de relever de 10 points le taux du PFU. Celui ci est aujourd’hui bien inférieur à ce qu’il était à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et au taux d’imposition maximal des revenus du travail. travail. En relevant le PFU de 10 points, on créerait davantage d’équité fiscale et on éviterait de priver la protection sociale de ressources lorsque les dividendes sont préférés aux salaires,

62 % des dividendes sont déclarés par 0,1 % des foyers fiscaux, soit 40 000 foyers, et 33 % par 0,01 % des foyers fiscaux, soit 4 000 d’entre eux. Ces proportions sont stables depuis 2018 et supérieures de 5 à 10 points aux niveaux constatés sur les années 2018 2017. Oui, la concentration des revenus mobiliers reste à un niveau très élevé, et c’est le résultat de votre politique ! La parole

mais seulement de l’évaporation, comme le souligne souvent notre collègue Éric Bocquet. En effet, rapport après rapport, étude après étude, cette décision apparaît

un ISF qui intégrerait un mécanisme novateur réservant les déductions fiscales aux investissements dans les entreprises écoresponsables, identifiées par l’attribution d’un label. Il est temps de réduire les inégalités, de réaligner notre politique fiscale sur les principes de justice sociale et de corriger les erreurs commises en 2017.

la mise en place d’un outil de justice climatique comprenant un système de bonus malus lié à l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers.

ce système de bonus malus, par la rénovation thermique de leur patrimoine immobilier, par l’abandon des actifs surconsommateurs d’énergie, comme les jets privés ou les yachts, ou par la réorientation de leurs investissements bancaires vers des projets plus durables et moins carbonés. Nous nous basons à cette fin sur la taxonomie du règlement 2020/852 du Parlement européen et

respectant cette démarche et de la réduire à 50 % dans le cas contraire, comme dans les pays scandinaves. Alors que 75 % des forêts en France sont des propriétés privées, notre conception exclusive du droit de propriété rend impraticable le principe, pourtant consacré

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par cet amendement, il est proposé d’encourager les ménages aisés à mettre en location des biens en sortant de l’assiette de l’IFI les logements concernés, sous condition de loyer et de ressources. Il pourrait être pertinent de renforcer la conditionnalité du dispositif en imposant un conventionnement de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Une telle mesure est complémentaire et cohérente avec l’alourdissement de la fiscalité sur les logements vacants et la politique de baisse des loyers. Elle permettrait, à court terme, de remettre sur le marché locatif plusieurs dizaines de milliers de logements,

Monsieur le ministre,

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

3,8 tonnes d’équivalent CO2, celle des 1 % les plus riches avoisine les 40 tonnes. Nous vous proposons de corriger cet écart considérable. La lutte contre la pollution et le changement climatique nécessite une action collective à tous les niveaux de la société en fonction des émissions de chacun. Les politiques publiques,

d’après l’âge de l’usufruitier éventuel. » Ce droit à restitution est pratiqué notamment dans le cas d’une donation par un parent à son enfant de la nue propriété d’un bien. Le donateur se réserve ainsi l’usufruit du bien et prévoit que cet usufruit sera reversé au profit, par exemple, de son conjoint plus jeune au jour de son décès. Ces usufruits sont dits successifs : le premier, actuel, porte sur la tête du donateur ; le second, éventuel, sur la tête du conjoint survivant. Un tel mode de calcul est pénalisant pour le nu propriétaire dès lors qu’au décès du premier usufruitier, le second usufruit s’ouvre au profit d’une personne plus jeune.

et premier usufruitier. Selon cette interprétation, l’amendement serait donc sans objet., la disposition proposée pourrait aboutir à intégrer à la succession du donateur décédé cette restitution, et donc à en faire bénéficier des héritiers n’ayant

Monsieur le ministre,

pour sauvegarder les édifices cultuels, qu’ils soient classés, inscrits ou non protégés,

Cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Patricia Schillinger, vise à prendre en compte la situation spécifique des édifices religieux des communes situées dans les départements de droit local d’Alsace et de Moselle, en portant le taux de la réduction d’impôts prévue par le code général des impôts de 66 % à 75 % pour les dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 dans le cadre de la collecte effectuée au profit de la Fondation du patrimoine

la souscription est de soutenir les communes dans le financement de la conservation de leur patrimoine religieux. L’instauration de cette souscription

l’avis du Gouvernement ? Quel est l’avis du Gouvernement ? La collecte nationale de dons au profit de la Fondation du patrimoine vise à financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux,

Comme l’a rappelé le rapporteur général, le dispositif est très utile pour nos communes, qui ont de plus en plus de mal à entretenir et à restaurer leur patrimoine religieux

intercommunalités qui se sont constituées en communes nouvelles. La plus grande de ces villes – ou de ces « villages », selon la nouvelle définition du Président de la République – était de 6 000 habitants.

une chose : quand on propose une idée, mieux vaut qu’elle soit bien pensée et bien cadrée ! Monsieur le ministre, la Président de la République a annoncé au mois de septembre le lancement de ce dispositif pour sauver le patrimoine religieux de nos villages.

Pour attirer ces dernières, il faudrait non seulement les exonérer de tout impôt, mais même appliquer cela à leurs salariés ! La Fédération

d’une fédération sportive pourraient ne pas payer d’impôts, contrairement aux autres citoyens ? Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. La parole est à M. le rapporteur

Fédération internationale de l’automobile, qui est reconnue par le CIO depuis 2012 et dont le siège est à Paris, Fédération internationale de football américain et, surtout,

Pé. Monsieur le président, monsieur le ministre,